Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons bientôt au terme de ce marathon budgétaire. Les missions qui nous occupent à présent sont assurément moins difficiles et moins débattues que d'autres, d'autant que leurs budgets sont relativement constants. qu'elles traduisent, elles aussi, certaines tendances de nos politiques publiques. Les montants annoncés de la mission « Pouvoirs publics » sont en légère hausse, pour répondre au contexte inflationniste. Ce constat vaut pour toutes les institutions, présidence de la République, Sénat et Assemblée nationale. C'est une bonne chose, même si nous pourrons toujours regretter des imprécisions dans les crédits demandés, en particulier lorsqu'il est question de dépenses de fonctionnement. J'observe qu'il est de plus en plus tenu compte de la performance énergétique des bâtiments- cela vaut aussi pour le palais du Luxembourg -, à l'heure de la lutte contre les passoires énergétiques ; nous y sommes vigilants. Quoi qu'il en soit, le budget de cette mission est relativement stable et sans vagues. Dans des périodes où certains croient qu'il faudrait tout renverser, tout bouleverser, dans la précipitation, et ce sans même avoir de véritable perspective, on ne se plaindra pas d'observer un peu de stabilité dans nos institutions.

sont en hausse, nonobstant les modifications de son périmètre ; la hausse principale va au renforcement des effectifs alloués à la cybersécurité et à la protection des données personnelles. C'est l'occasion pour moi de dire mon inquiétude sur tous ces sujets. Certes, je suis d'une génération qui n'est pas toujours très au fait des dernières avancées technologiques : il est vrai que je préfère le papier aux écrans, le livre aux tablettes et le stylo à l'index. Toujours est-il qu'avec le développement de ces nouveaux outils je comprends bien qu'il faille faire face à une hausse constante des cyberattaques, lesquelles touchent directement les intérêts de l'État et de notre Nation.

salue notamment un nouveau renforcement des moyens attribués à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Je conclurai brièvement en abordant la question du contentieux administratif. Nous ne pouvons que nous féliciter de la hausse des crédits dans un contexte de croissance continue dudit contentieux. Nous le disions lors de l'examen de la mission « Justice », ces phénomènes d'inflation et d'engorgement des juridictions doivent être endigués ; espérons que ces moyens y participeront. recommandations de notre rapporteur spécial Christian Bilhac, qui invite notamment le Conseil d'État à se saisir pleinement de son rôle de gestionnaire des juridictions administratives. Il n'en demeure pas moins que notre groupe votera en faveur de l'ensemble de ces crédits.

Gouvernement ». Les crédits de la mission « Pouvoirs publics » connaissent une faible progression, de l'ordre de 2,76 %, par rapport à 2022. Cette hausse très modérée résulte principalement du contexte inflationniste et de la volonté des pouvoirs publics de maintenir un certain niveau d'investissement. À cet égard, je tiens à rappeler, pour les saluer, les efforts budgétaires consentis par les différentes institutions depuis une dizaine d'années. d'années. La mission « Conseil et contrôle de l'État » rassemble notamment les crédits alloués aux juridictions administratives et financières. Son objet est de donner à ces institutions indispensables à notre démocratie les moyens de leurs attributions. Une hausse de ses crédits de l'ordre de 8,5 % est prévue est la bienvenue, car il est fondamental que l'État octroie des dotations suffisantes à son propre contrôle. La mission « Direction de l'action du Gouvernement », quant à elle, voit ses crédits augmenter de 3,5 % en crédits de paiement et de 9 % en autorisations d'engagement. Cette hausse traduit notamment la priorité donnée par le Gouvernement à la protection des données et à la lutte contre la cybercriminalité, dans un contexte de cyberattaques frappant aussi bien les collectivités territoriales et l'État que les entreprises et les centres hospitaliers. Nous gardons tous en mémoire le piratage informatique qui a visé l'hôpital de Corbeil-Essonnes en août dernier. Aussi, je souhaite souligner le renforcement de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui verront leurs effectifs augmenter. parallèle, la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique verra également ses moyens s'accroître, en réponse à l'extension de ses compétences à de nouveaux acteurs du numérique, tels que les réseaux sociaux, les plateformes et les sites de partage de vidéos. Je me réjouis donc du renforcement substantiel des moyens destinés à la cybersécurité, car il s'agit d'un enjeu crucial face à une menace cyber qui ne cesse de croître. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ces crédits, quoique très hétérogènes, sont tous essentiels au bon fonctionnement de notre État de droit. Ils tendent à assurer aux pouvoirs publics, aux organes chargés de leur contrôle, ainsi qu'aux autorités indépendantes qui veillent au respect des libertés individuelles, les moyens nécessaires à leur action. Aussi, le groupe Les Indépendants - République et Territoires votera les crédits de ces trois missions.

de la Cnil et de l'Arcom augmentent, ce qui est positif ; mais ils demeurent en deçà des besoins. Quant aux crédits prévus pour le Défenseur des droits, ils nous semblent bien trop faibles. Concernant les enjeux de santé publique, nous nous étonnons de la faible hausse des crédits accordés à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives alors même que le ministre de la santé entend faire de la prévention un axe fort de politique publique. Concernant la protection de notre démocratie et la diffusion des idées, nous nous inquiétons que les crédits alloués aux fondations politiques soient si bas. En encourageant ainsi leur recherche de financements privés, nous prenons le risque d'affecter leur fonctionnement.

mais ces mesures ne doivent pas être un joli affichage pastillé de vert dans votre budget ... Le Haut Conseil pour le climat est devenu un acteur indispensable du débat public en matière d'action climatique.

dont il fait l'objet de la part du Gouvernement, du Parlement, des collectivités territoriales, mais également de la presse et de la société civile. Nous suivrons donc très attentivement l'évolution de son budget et veillerons à l'effectivité de la hausse des effectifs prévue. Le secrétariat général à la planification écologique que vous proposez de créer bénéficiera, quant à lui, de 15 ETP et de 500 000 euros de budget. Au regard de la tâche que représente la planification écologique

Alors que les risques environnementaux et sociaux s'enchevêtrent chaque jour davantage, compte tenu de la montée en puissance des effets du réchauffement climatique et, plus largement, des impacts de l'être humain sur l'environnement, nous avons besoin de mesures concrètes, prévues sur le long terme, prises dans une vue d'ensemble, pour assurer une réelle transition écologique. nous proposons au Gouvernement la création d'un ministère des risques. La situation mondiale nous montre que nous devons anticiper tous les risques, qui finissent par se recouper : crise sanitaire mondialisée, qui affecte notre économie

afin de les prévenir ou d'y répondre plus efficacement. Je conclurai en rappelant que ce budget, dans son ensemble, demeure insuffisant pour faire face aux enjeux écologiques majeurs qui nous attendent ; il trahit un manque de vision globale et à long terme sur le sujet de la part du Gouvernement. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. La

Permettez-moi tout d'abord de saluer les efforts budgétaires consentis au cours des dernières années par les institutions relevant de la mission « Pouvoirs publics ». Au regard de la poussée inflationniste actuelle, la hausse des crédits demandés à leur profit pour 2023 apparaît tout à fait justifiée. Pour ce qui concerne la présidence de la République, l'augmentation des crédits de fonctionnement est parfaitement légitime, étant donné la nécessité de garantir la sécurité du chef de l'État et des personnels de l'Élysée. qui est de la mission « Conseil et contrôle de l'État », la poursuite du renforcement des moyens alloués aux juridictions administratives est bienvenue, eu égard à la forte progression de l'activité contentieuse. La création de 202 nouveaux emplois entre 2023 et 2027 devrait notamment permettre aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel de réduire leurs stocks d'affaires en attente. Les préoccupations soulevées par le rapporteur pour avis Benarroche méritent, selon moi, d'être prises en considération. Il faudra en effet veiller à ce que la nouvelle obligation de mobilité statutaire ne nuise pas à la gestion prévisionnelle des effectifs. Par ailleurs, je me réjouis de constater que le renforcement des moyens de la Cour nationale du droit Malgré une augmentation très forte du nombre de recours, la cour a réussi à réduire ses délais de jugement, ainsi que son stock d'affaires en attente. Il reste à espérer que les moyens dont elle dispose lui permettront d'atteindre les objectifs fixés par la réforme de l'asile.

À l'instar du rapporteur pour avis susnommé, je pense qu'il sera nécessaire de veiller à ce que la mise en oeuvre de cette réforme ne nuise pas aux missions traditionnelles des CRTC. Un autre motif de satisfaction est l'ouverture des crédits nécessaires à la mise en place de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement, dont le secrétariat général sera assuré par la Cour des comptes. Je rappelle que le groupe RDPI a pris une part active à la définition des contours de cette commission, dont la création vise à répondre à la demande accrue de redevabilité de l'aide publique au aux crédits de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ». Je tiens avant tout à souligner la décision du Gouvernement de poursuivre le renforcement des moyens alloués à l'Anssi. Ce nouvel effort budgétaire est indispensable au regard de l'accroissement de la menace cyber et de l'impérieuse nécessité de prévenir les cyberattaques pouvant causer des dommages physiques. Les attaques qui ont récemment frappé des centres hospitaliers et des collectivités territoriales montrent combien il est urgent de renforcer la lutte contre la cybercriminalité. À cet égard, il convient de se féliciter de l'ouverture à Rennes d'une nouvelle antenne de l'Anssi, qui viendra parachever la mise en place, dans la capitale bretonne, d'un pôle de compétence en cyberdéfense unique en Europe. La construction d'un véritable écosystème cyber permettra à la France d'être mieux armée pour affronter les trois grandes menaces que sont la menace criminelle, l'espionnage et la menace militaire. La lutte contre la désinformation est un autre défi majeur, qui justifie le renforcement des moyens alloués au Viginum et à l'Arcom. Enfin, réjouissons-nous également de la mise en place du secrétariat général à la planification écologique, qui trouve sa traduction budgétaire dans ce projet de loi de finances. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le groupe RDPI votera les crédits de ces trois missions.

les trois missions dont nous étudions les crédits aujourd'hui bénéficient toutes d'une hausse des moyens alloués. S'il convient de souligner cette augmentation, quelques remarques s'imposent par évoquer la mission « Pouvoirs publics ». À l'exception du Conseil constitutionnel, qui voit ses moyens diminuer de 16,7 %, et de la Cour de justice de la République, dont les crédits sont stables, toutes les dotations sollicitées sont à la hausse, et ce pour des raisons qui tiennent essentiellement à l'inflation et aux surcoûts liés à la revalorisation du point d'indice de la fonction publique. Ce contexte inflationniste incontestable ne saurait pour autant tout expliquer. Ainsi, pour la présidence de la République, les dépenses de fonctionnement sont attendues en hausse de 12,5 %, soit plus du double du niveau de l'inflation. Comme l'a expliqué Jean-Pierre Sueur, le « recalibrage [ ...] permettant de faire face aux coûts de gestion courante », censé à lui seul justifier cette hausse, manque pour le moins de précision. Les deux assemblées voient également leur budget augmenter. Celui des chaînes parlementaires se maintient, ce qui permet de faire face à l'augmentation des coûts de diffusion. La mission « Conseil et contrôle de l'État », aux budgets des juridictions administratives, des juridictions financières et du Conseil économique, social et environnemental, connaît elle aussi une hausse notable de ses crédits. Les dépenses de personnel augmentent de 9 %, essentiellement pour renforcer les effectifs du Conseil d'État et des juridictions administratives. vu de l'augmentation du contentieux devant les juridictions administratives, des moyens supplémentaires sont bel et bien indispensables pour tenter de donner des réponses aux justiciables dans des délais raisonnables. Néanmoins, ces délais restent une source d'inquiétude, d'autant que le stock s'est de nouveau accru. Les mêmes inquiétudes se portent sur la Cour nationale du droit d'asile ; le Gouvernement estime que les créations d'emplois des années précédentes doivent permettre de tenir l'objectif d'un délai et ce malgré le nombre croissant de recours. Par ailleurs, il conviendra de veiller à ce que la généralisation des téléprocédures, présentée comme un moyen de rationalisation du travail des agents de greffe et de facilitation de l'instruction par les magistrats, ne nuise pas à la qualité des décisions rendues et à l'accès au droit des administrés. Les recommandations du Conseil d'État- promouvoir le règlement amiable des litiges, notamment par la voie de la médiation -semblent également pertinentes pour limiter l'augmentation du contentieux. Enfin, la mission « Direction de l'action du Gouvernement » regroupe deux programmes de natures assez différentes, qu'il convient donc d'évoquer distinctement. En raison de la suppression du programme destiné à couvrir les dépenses liées à la présidence du Conseil de l'Union européenne, exercée par la France au premier semestre 2022, les crédits destinés à cette mission paraissent en baisse

Dans un contexte de hausse inquiétante de la cybercriminalité, frappant aussi bien l'État que les collectivités territoriales, les hôpitaux que l'ensemble des services publics, ce renforcement des moyens destinés à la lutte contre ce fléau est une très bonne chose. Ainsi, les renforts en personnel au bénéfice du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, et principalement pour l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, sont à saluer. Si l'on peut noter avec satisfaction la modération des crédits alloués au service d'information du Gouvernement (SIG), son cas ne laisse pas malgré tout de nous interpeller, car, je le rappelle, la Cour des comptes pointe chaque année un niveau de dépenses nettement supérieur au budget voté. Les dépenses du SIG mériteraient d'être mieux calibrées afin que l'on ne puisse pas remettre en question la sincérité des comptes. À ce propos, une information plus claire- et même une information tout court -ne saurait nuire concernant l'activité du Haut-Commissariat au plan. Visiblement, ce ne sera pas non plus pour cette année Fort heureusement, il est aussi des sujets sur lesquels nous disposons d'éléments nous permettant d'apprécier l'évolution de certains services et institutions. Il convient ainsi de saluer le travail effectué au sein de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la Mildeca, dont les moyens sont cette année réajustés, après une diminution continue depuis 2019. Plus globalement, le programme 308, « Protection des droits et libertés », connaît lui aussi une revalorisation de ses moyens.

Si ces deux institutions concentrent l'essentiel des effectifs, les besoins humains et financiers des autres autorités indépendantes méritent d'être consolidés.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la mission « Pouvoirs publics » comprend les crédits de la présidence de la République, du Conseil constitutionnel, de la Cour de justice de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la chaîne parlementaire, notamment.

devait soi-disant « conforter la place et le rôle de la troisième assemblée au sein du paysage institutionnel de la République ».

Le président Macron, contraint d'alimenter la chose qu'il a lui-même créée, a annoncé le 13 septembre dernier le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie, dont le pilotage a été confié, je

Pour l'année 2023, le Cese dispose d'une enveloppe budgétaire de 4,2 millions d'euros, je l'ai dit, entièrement fléchée vers la participation citoyenne. L'institution gère directement ces crédits, contrairement aux années précédentes, où ils devaient être débloqués par le Gouvernement. Le rapporteur spécial a donc bien raison d'indiquer qu'il entend être attentif à l'utilisation de ces crédits, notamment du point de vue de la sincérité budgétaire. Comme l'on pouvait s'y attendre, en juin 2022, une direction de la participation citoyenne a été créée au sein du Cese.

Madame la présidente,

qui ont produit, cette année encore, un travail d'analyse d'une grande qualité sur ces crédits. Ces trois missions budgétaires fixent les dotations d'institutions d'une grande diversité, qui ont pour point commun de contribuer de manière déterminante au respect des principes fondamentaux de notre démocratie et au bon fonctionnement de l'État. Permettez-moi d'évoquer, en premier lieu, la mission « Pouvoirs publics », dont l'enveloppe globale est cette année de 1,08 milliard d'euros, en légère hausse de 2,8 %. Cette mission présente une certaine singularité, car elle regroupe le budget de plusieurs institutions de nature constitutionnelle, qui jouissent d'une autonomie financière sur le fondement de la séparation des pouvoirs. Comme le veut l'usage, je m'abstiendrai de toute observation sur le budget du Sénat et de l'Assemblée nationale, fixés par la commission commune compétente en la matière. Pour ce qui concerne le Conseil constitutionnel, si l'on neutralise l'effet d'une baisse optique liée aux dépenses nécessaires au contrôle et au contentieux des élections en 2022, sa dotation est stable, à 13,3 millions d'euros, et lui permettra d'exercer ses missions dans de bonnes conditions, comme l'a rappelé M. le questeur Sueur. La Cour de justice de la République disposera quant à elle d'un budget reconduit à 980 000 euros pour assurer le traitement des requêtes visant les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions

dans cette période de crise, et de mener à bien des investissements indispensables à la modernisation des emprises et à la sécurisation de la présidence, comme l'a très justement souligné le rapporteur spécial M. Arnaud.

et financières d'exercer pleinement leurs missions, qui sont au coeur des attributions régaliennes de l'État, comme l'indiquait M. Bilhac dans son rapport. Pour ce qui est du Conseil d'État et des juridictions financières, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit la création de 41 emplois supplémentaires, dont 25 magistrats, destinés à renforcer les juridictions aux fins de faire face à l'augmentation du nombre de recours. Je sais, monsieur Benarroche, que vous êtes attentif à cette question des ressources humaines des juridictions. Cet effort est indispensable pour assurer la maîtrise des délais de jugement, qui demeure une préoccupation majeure pour la juridiction administrative. La Cour des comptes et les juridictions financières verront également leurs crédits progresser sous l'effet de la hausse du point d'indice, de revalorisations liées à la réforme de la haute fonction publique et de la mise en place de la Commission d'évaluation de l'aide publique au développement, créée par la loi de

Enfin, la dotation budgétaire du Conseil économique, social et environnemental est stable, à 45 millions d'euros. En cohérence avec les principes de la réforme organique du 15 janvier 2021, le Cese,

j'évoquerai la mission « Direction de l'action du Gouvernement », consacrée à la coordination du travail gouvernemental, ainsi qu'à plusieurs autorités indépendantes essentielles à la protection des droits et libertés. Les crédits des deux programmes de la mission augmentent de 8 %, pour une enveloppe totale de 926 millions d'euros. Les crédits du programme « Coordination du travail gouvernemental » sont en hausse sous l'effet d'un schéma d'emplois de 129 emplois supplémentaires, dont 95 pour le SGDSN pour le SGDSN et les organismes rattachés, qui doivent faire face à des enjeux de cybersécurité toujours plus importants. Comme l'ont rappelé MM. Leconte, Cadic et Vallet dans leurs travaux respectifs, il est essentiel de renforcer les moyens des services de l'État pour faire face à ces menaces croissantes.

Des créations d'emplois accompagneront la mise en place du secrétariat général à la planification écologique et du Conseil national de la refondation. Je sais, monsieur Parigi, que vous suivrez avec attention l'activité du SGPE, qui doit jouer un rôle déterminant déterminant pour la transition écologique de notre pays. Enfin, la Diese sera renforcée pour mettre en oeuvre la réforme engagée depuis 2021 et promouvoir une haute fonction publique plus forte, plus ouverte et plus mobile au service de l'intérêt général. Le programme « Protection des droits et des libertés » bénéficie également d'emplois supplémentaires qui doivent permettre aux autorités indépendantes qui lui sont rattachées d'exercer au mieux leurs prérogatives.

territoriaux et de revaloriser leur indemnité. Enfin, j'évoquerai les crédits de la direction de l'information légale et administrative (Dila), dont le budget devrait être excédentaire pour l'année 2023. La Dila poursuivra la transformation de son fonctionnement et l'actualisation de ses outils numériques, qui contribuent au quotidien à l'information des citoyens et à la connaissance des politiques publiques. Je conclurai, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, en vous demandant d'adopter les crédits de ces trois missions et du budget annexe. Mes chers

Sous prétexte de la suppression du contrôle juridictionnel des comptables publics, le projet de loi de finances pour 2023 supprime toute mention du contrôle des comptes dans les indicateurs de performance. Par ailleurs, pour mesurer l'objectif « Sanctionner les irrégularités et la mauvaise gestion », il ne prévoit qu'un seul indicateur, relatif aux délais de jugement de la chambre du contentieux de la Cour des comptes, alors que le premier objectif devrait être d'alimenter cette nouvelle chambre en dossiers, les déférés qui arrivent des cours régionales.

indicateur documenterait le nombre de contrôles des comptes et de la gestion menés auprès des collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants. On connaît, en effet, l'importance de ces contrôles pour des communes qui ne disposent pas des moyens d'ingénierie des grandes collectivités. indicateur documenterait les effets sur les comptes des travaux de contrôle des comptes et de la gestion en retraçant le nombre de recommandations faites en matière de fiabilité et de qualité des comptes, comme cela existe déjà pour les travaux de certification. indicateur a trait au nombre de déférés à la chambre du contentieux effectués par la Cour des comptes et par les chambres régionales et territoriales des comptes. Enfin, afin de valoriser les nouvelles missions des chambres régionales des comptes créées par la loi 3DS, cet amendement tend à introduire un quatrième indicateur relatif au nombre de rapports établis par celles-ci en matière d'évaluation des politiques publiques territoriales et d'avis sur les les conséquences de projets d'investissements exceptionnels. Les deux derniers indicateurs présentés concernent des dispositions qui entrent en vigueur en 2023 ; il convient donc qu'ils fassent l'objet de prévisions prudentes pour prendre en compte le nécessaire rodage de ces nouvelles procédures. L'adoption de cet amendement aurait pour effet de rétablir dans le projet de loi de finances pour 2023

donc pour le moins précoce d'adapter les indicateurs. D'ailleurs, la Cour des comptes nous a informés que, dès 2024, il y aurait une évolution de ces indicateurs, et que nous pouvions d'ores et

monsieur le ministre,

aux fondations politiques. Cette augmentation du budget doit aussi permettre à ces structures de limiter leur recherche de financements privés afin de restreindre les conséquences sur leur fonctionnement interne. En mai 2022, Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, a indiqué qu'il envisageait d'inscrire les au registre des lobbies, au regard du poids parfois très important des financements privés dans leur fonctionnement, poids qui n'est pas sans incidence sur le choix des sujets étudiés et sur leur approche. En résumé, cette hausse des moyens alloués aux fondations politiques, qui sont

D'une part, il est important de donner quelques moyens complémentaires au Défenseur des droits, compte tenu de l'élargissement de son périmètre d'intervention à la défense des lanceurs d'alerte loi de mars 2022, mais aussi de l'augmentation du nombre de réclamations, qui sont de plus en plus difficiles à traiter. Il est important, en particulier, de renforcer les pôles régionaux du Défenseur des droits, raison pour laquelle nous proposons la création de 3 ETP.

considérons qu'il ne sert à rien et qu'il constitue un doublon avec le Conseil économique, social et environnemental, pour doter un peu davantage le Défenseur des droits, qui en a bien besoin. Quel est l'avis de la commission ?

brouillard insusceptible de faire avancer les choses. Cela a été dit par tant de responsables de toute nature dans le monde social et politique que je ne comprends pas que vous vous obstiniez à donner un semblant de crédibilité à cet appareil- ce dispositif, cette instance, que sais-je -qui n'en a aucune. Cet amendement est donc vraiment très justifié, et M. Leconte a eu grandement raison de nous le présenter

bonne nouvelle, il ne coûte que 1 euro ! Ce n'est pas rien ! Cet amendement d'appel a pour objet d'encourager le Gouvernement à agir de façon plus globale et transversale face aux risques mondiaux actuels et à venir, par la création d'un ministère des risques. tous les autres ... Nous faisons face à de nombreux risques interconnectés, que nous devons anticiper dans nos politiques publiques. Ces risques sont environnementaux, sociaux, sanitaires, démocratiques ; nous devons les prévenir et apprendre à mieux y parer. Je parle de la crise du covid-19, qui a démontré la faiblesse de nos réponses sanitaires dans une économie mondialisée capitaliste. Je parle du réchauffement climatique, qui est déjà là, 2022 étant l'année la plus chaude jamais mesurée en France et de terribles incendies ayant défiguré le pays cet été.

parle aussi de la guerre en Ukraine et de ses répercussions sur le coût de l'énergie et sur notre pouvoir d'achat, ou encore des dangers réels de bombardements de centrales nucléaires. Tous ces faits témoignent de ce que les risques environnementaux et sociaux s'enchevêtrent

et, de manière récurrente, voire récursive, d'encourager le Gouvernement à intensifier les efforts budgétaires en faveur du rattrapage des écarts forts et persistants qui demeurent entre les territoires d'outre-mer et la France métropolitaine dans les domaines socio-économiques.

Si la progression des crédits du programme 138 reste relative et tend à être neutralisée par l'inflation, cette hausse est incontestable sur le programme 123, du fait du développement de dispositifs de soutien exceptionnel aux collectivités, avec une augmentation de 7,19 % en autorisations Ces efforts sont importants, mais la tâche reste immense au lendemain de la crise sanitaire ayant touché brutalement les économies de nos territoires éloignés. Globalement, et de manière plus marquée dans certains territoires, les écarts avec la métropole ont eu tendance à s'accroître, en dépit des efforts de tous pour juguler la crise. Ainsi, le PIB par habitant enregistre, en moyenne, une légère diminution en outre-mer entre 2019 et 2021, alors qu'il enregistre une hausse de plus de 5 % en métropole. En Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, le PIB par habitant a diminué entre 2019 et 2021. Dans les autres territoires d'outre-mer, il enregistre une progression comprise entre 1,93 % et 3,78 %, contre 5,22 % en métropole. Les évolutions démographiques sont contrastées entre les différents bassins océaniques ; elles font naître des besoins nouveaux qui diffèrent selon le profil de la pyramide des âges, tantôt jeune et croissante- en Guyane, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française -, tantôt en baisse et vieillissante, notamment dans les Antilles.

la Guyane et la Polynésie française étant plus durement touchées que la métropole. Les habitants de nos collectivités ultramarines sont bien affectés par l'inflation, qui enregistre une hausse notable malgré l'existence du bouclier qualité-prix mis en place en 2012. cette inflation s'ajoute à un coût de la vie déjà structurellement supérieur dans les territoires d'outre-mer, renchérissant encore l'approvisionnement des ménages, des entreprises et des collectivités ultramarines. Si des annonces ont pu être faites par le Gouvernement au banc de l'Assemblée nationale, nous restons attentifs à toute initiative visant à limiter l'inflation en outre-mer et à protéger le pouvoir d'achat des citoyens français ultramarins, en particulier sur le plan des produits alimentaires. Il résulte de ce contexte économique que la situation financière des collectivités d'outre-mer se détériore. Certaines d'entre elles n'ont plus les moyens de leurs investissements, pourtant si nécessaires. Cette dégradation structurelle de leur situation financière explique d'ailleurs en partie les problèmes de sous-consommation régulièrement constatés sur la mission. de soutenir les collectivités ultramarines ; ce soutien doit même être renforcé en cette période de crise économique. Face aux écarts de développement et à une pauvreté qui peine à se résorber, le contexte de tension sociale a conduit à faire entendre plus fortement, en mai 2022, la voix des élus des outre-mer. Si cet Si cet appel au changement des politiques d'aide au développement dans les territoires d'outre-mer a donc été entendu, la réponse attendue ne saurait se limiter à sa seule dimension financière. Sur ce plan particulier, néanmoins, l'effort doit certes passer par les crédits de la mission- c'est le cas -, mais également par les crédits des autres missions du budget de l'État et par les dépenses fiscales. les dépenses fiscales rattachées à la mission enregistrent, en 2023, une nouvelle hausse : elles passent de 6,916 milliards d'euros à 7,090 milliards d'euros. Nous saluons d'ailleurs la prolongation jusqu'en 2029 de nombreux dispositifs fiscaux qui devaient s'éteindre en 2025. Le Sénat

et que d'autres sont prévues pour 2023. Ces évaluations demeurent un exercice complexe, à la fiabilité relative, mais elles représentent un préalable nécessaire à une réflexion plus large sur les dépenses fiscales et à un maintien légitimé des dispositifs de défiscalisation. De surcroît, en complément des dépenses fiscales, les territoires d'outre-mer bénéficient de crédits en provenance d'autres programmes du budget général, qui sont retracés dans le document de politique transversale « outre-mer ». Ces crédits proviennent de 101 programmes budgétaires relevant de 32 missions, dont 48 programmes ayant trait à l'emploi, à l'égalité des chances, aux conditions de vie, à l'aménagement durable, aux dotations aux collectivités territoriales

Ces taux sont décevants et doivent nous conduire, à l'avenir, à nous montrer vigilants, notamment pour éviter des redéploiements en cas d'absence de consommation. Toutefois, les crédits du plan de relance ont eu un effet de levier important sur le financement des collectivités ils ont permis de financer des projets indispensables aux territoires d'outre-mer et de renforcer des dispositifs existants, comme les contrats de convergence ou la ligne budgétaire unique (LBU). À cet égard, il est important de souligner que, lorsqu'ils ont été orientés sur des dispositifs existants, les crédits ont été intégralement consommés.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la mission « Outre-mer » a pour principal objectif le rattrapage des écarts persistants entre l'outre-mer et la métropole et la convergence des niveaux de vie dans le domaine socio-économique. Ces crédits sont essentiels pour les territoires ultramarins en ce qu'ils représentent des aides exceptionnelles ou complémentaires aux dotations de fonctionnement et d'investissement classiques allouées à l'ensemble des collectivités.

Ces nouveaux crédits permettront notamment de financer le renforcement de l'assistance technique aux collectivités, le développement de l'alimentation en eau potable en Guadeloupe, le soutien aux dispositifs de lutte contre le changement climatique dans le Pacifique, en matière de diversification agricole et, enfin, la réforme de la fonction publique territoriale dans les îles Wallis et Futuna. Si l'on peut se réjouir de ces augmentations de crédits, d'autres points plus préoccupants méritent d'être soulignés. Les crédits ouverts au titre de la ligne budgétaire unique ne permettent pas de répondre aux besoins dans ce domaine, notamment concernant la résorption de l'habitat insalubre. C'est pourquoi nous vous proposerons un amendement visant à augmenter de 4 millions d'euros les crédits alloués à cette résorption. Cette ouverture se justifie d'autant plus que les crédits ouverts les dernières années ont été intégralement consommés.

Cependant, dans un contexte économique qui accentue la dégradation de la situation financière des collectivités d'outre-mer, nous estimons que ce dispositif doit être encore renforcé pour s'étendre à un nombre plus important de collectivités.

Toutefois, les crédits alloués aux exonérations de charges enregistrent, à périmètre constant, une hausse de plus de 202,7 millions d'euros. Dans un contexte économique incertain, il est délicat, à ce stade, d'établir une prévision fine

et par le déploiement dans tous les territoires du SMA 2025+, qui a notamment pour objectif d'ouvrir le service militaire adapté à de nouveaux publics. Ce dispositif a démontré son efficacité, et son extension à des mineurs et à des mères célibataires permettra, sans aucun doute, une meilleure professionnalisation et une meilleure intégration de ces personnes. Nous devrons toutefois être vigilants sur les taux d'insertion qui seront enregistrés ces prochaines années, dans un contexte économique difficile. Enfin, les crédits destinés au financement de l'économie, c'est-à-dire les microcrédits, l'aide au fret et le prêt de développement outre-mer, restent stables, à 24 millions d'euros. Cette stabilité, bien que louable, pourrait cependant se révéler insuffisante pour couvrir les besoins réels en 2023. En effet, dans le contexte économique actuel, la situation des entreprises

Il reste toutefois beaucoup à faire et nous devons oeuvrer de concert pour une consommation accrue de ces crédits. Je pense sincèrement que les Corom sont une des solutions pour améliorer la situation financière financière des collectivités, leur capacité à investir et le niveau de consommation des crédits de la mission. Malgré les réserves évoquées, nous vous proposerons de voter les crédits de la mission « Outre-mer

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires économiques a choisi d'émettre un avis favorable sur l'adoption des crédits de la mission « Outre-mer » pour 2023, non sans réserves ni recommandations. Non sans réserves, dis-je, car, après analyse, les augmentations de crédits sont trop souvent modestes, ne couvrant pas même l'inflation prévue pour 2023

Ma première observation porte sur le logement. Le constat demeure inchangé d'année en année, celui d'un manque cruel de constructions comme de rénovations. Pour l'année 2021, ce sont 3 036 logements locatifs sociaux et très sociaux qui ont été livrés, alors que le besoin annuel est estimé à plus de 8 000. De même, 1 628 réhabilitations de logements sociaux ont été menées à leur terme, en dépit des financements importants du plan de relance. Concernant la lutte contre l'habitat insalubre, les crédits de 2022 sont reconduits, alors même que les besoins sont immenses.

Je souhaite également insister, dans la continuité des travaux menés par la délégation aux outre-mer, sur la nécessité d'organiser des assises de la construction, en préalable à l'établissement d'un troisième plan Logement Ma seconde observation a trait à la formation au sens large. Je tiens à souligner la nouvelle montée en puissance du service militaire adapté, lequel, s'il ne saurait constituer la seule réponse aux maux de notre jeunesse, reste un outil puissant d'insertion socio-économique.

Je m'étonne toujours que les territoires ultramarins, forts de leurs 2,8 millions d'habitants, ne disposent d'aucune école de commerce, école d'ingénieur ou institut Pourquoi les jeunes Ultramarins devraient-ils toujours aller étudier dans l'Hexagone ? Il est temps d'ouvrir une réflexion par bassin géographique sur l'offre d'enseignement supérieur présente en outre-mer. S'il est positif que les jeunes souhaitant étudier à Paris puissent le faire dans de bonnes conditions, pourquoi ne pas imaginer, demain, que de jeunes hexagonaux viennent suivre une formation d'excellence dans un territoire ultramarin ? Si l'on souhaite créer de la valeur sur place, conformément à votre souhait, monsieur le ministre, il faut s'en donner les moyens.

je vous remercie Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, si elle ne s'est pas opposée à l'adoption des crédits de la mission « Outre-mer » inscrits dans le projet de loi de finances pour 2023, la commission des lois a émis des réserves sur trois points qu'il m'appartient aujourd'hui de vous présenter. Tout d'abord, le contexte dans lequel s'inscrit l'examen du projet de loi de finances pour 2023 n'est pas neutre : la persistance de la crise énergétique et les tensions inflationnistes exacerbent les problématiques de la vie chère et les difficultés propres aux territoires ultramarins. Pourtant, force a été de constater le défaut d'adaptation des mesures nationales aux spécificités des collectivités et des entreprises ultramarines.

dans les dispositifs proposés pour compenser en 2023 la hausse des prix de l'énergie pour les collectivités, les ménages et les entreprises. Nous resterons vigilants quant au suivi et à l'application territorialisée de ces mesures dans nos outre-mer. Par ailleurs, la principale problématique à laquelle est confrontée la mission « Outre-mer » est celle de la sous-exécution chronique des crédits votés, bien que des efforts aient récemment été entrepris en la matière. Cet état de fait n'est acceptable pour les citoyens, qui ne comprennent pas que les crédits ne parviennent pas jusqu'à eux ; ni pour les collectivités ultramarines- leur situation et les défis auxquels elles font face imposent une politique particulièrement volontariste et pleinement engagée de l'État ; ni pour nous, législateurs, qui voyons notre intention contrariée par la sous-consommation de crédits pourtant votés, parfois même obtenus de haute lutte, dans l'hémicycle. L'accompagnement des collectivités ultramarines

passe par les contrats de convergence et de transformation, qui doivent impérativement être consommés et améliorés pour l'avenir, par le fonds exceptionnel d'investissement (FEI), mais également par le dispositif des Corom, que nous vous proposerons de renforcer. Le budget pour 2023 démontre ainsi une nouvelle fois que les problèmes d'ingénierie dans nos collectivités méritent une réponse adaptée et volontariste ; comme je l'ai annoncé en commission des lois, je déposerai prochainement une proposition de loi pour y remédier. Au bénéfice de ces observations, la commission des lois a donné un avis favorable sur l'adoption de ces crédits.

Dans cet exercice récurrent, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, les parlementaires vous diront rarement merci, monsieur le ministre ; ils préféreront vous interpeller sur les attentes de nos concitoyens ou sur les manquements criants

Notre éloignement engendre des surcoûts permanents causés par la faiblesse concurrentielle et une situation oligopolistique consolidée d'année en année. Concernant l'emploi, monsieur le ministre, on vous renverra aux chiffres du chômage plutôt que de rappeler l'augmentation des crédits du FEI ou le travail salutaire du Non, nous ne sommes pourtant pas des ingrats ! S'il leur arrive de susciter de l'agacement chez nos compatriotes de l'Hexagone, qui estiment que l'on pleure facilement au soleil, il est aussi vrai que les Domiens se sentent incompris.

perspective, nous devons penser en « mériens » et non pas en terriens. Cela n'est pas toujours simple, alors que l'État exerce une compétence exclusive sur les taxes et sur le domaine de la pêche et que l'Union européenne détient toutes les compétences sur les eaux communautaires, sans qu'aucune collectivité ultramarine y soit associée.

celui de la grande capitale parisienne. Chez nous, c'est la France, mais qu'en est-il vraiment, entre surcoûts de fret, octroi de mer, frais de poste exorbitants et droits de douane particuliers ? Chez nous, c'est la France, mais de ceux qui sont partis sans espoir de retour en famille, de retour au pays ? Non, nos compatriotes ne sont pas des ingrats, mais une large majorité d'entre eux a exprimé son mal-être et son malaise au travers de votes extrêmes. Qu'ont-ils voulu dire ? Ce que nous savons déjà : notre modèle économique monopolistique fondé sur des échanges commerciaux exclusifs entre la France et l'Europe n'est plus viable. Un cycle se termine. Ce modèle a permis des progrès évidents dans le monde d'avant, mais il a creusé des inégalités et suscité des frustrations. Quand bien même la République reste présente lors de chaque crise-

Payer moins cher leur électricité et utiliser l'énergie radiative du soleil. Pour cela, l'aide à l'investissement dans les énergies renouvelables est nécessaire ; à défaut, comment parvenir à l'autonomie énergétique ?

Tout simplement que nous agissions pour qu'ils vivent mieux, pour faire rimer « ultramarin » avec « ultra-humain ». Je vous demande donc de prendre en compte les différents amendements qui seront défendus par mes collègues et par moi-même, dont celui qui vise à augmenter les crédits alloués à la lutte contre les violences intrafamiliales dans les outre-mer. Un signal de votre ministère serait apprécié,

cette mission était de répondre aux préoccupations du quotidien, en portant une attention particulière aux sujets environnementaux. Je tiens tout d'abord à vous encourager dans cette volonté de réduire les inégalités entre tous les territoires, une tâche difficile dans un contexte inflationniste marqué par la menace d'une crise énergétique majeure. ajoutent les problématiques sécuritaires, l'immigration, l'insuffisance du pouvoir d'achat aggravée par la vie chère, le chômage de masse ou encore les conséquences de la crise sanitaire. Toutes ces crises rendent le quotidien de nos compatriotes ultramarins souvent insupportable.

Nous ne pouvons examiner les crédits de la mission « Outre-mer » sans aborder des sujets plus larges, comme la question sécuritaire à Mayotte. Depuis plusieurs jours, une escalade de violence secoue Mamoudzou, où des affrontements entre jeunes de quartiers rivaux ont fait un mort, un homme de 20 ans tué à la machette. À cela s'ajoute l'attaque sans compter le nombre de blessés qui ne cesse d'augmenter. Comme l'ont rappelé nos collègues la députée Estelle Youssouffa et le sénateur Thani Mohamed Soilihi, ce phénomène d'extrême violence ne date pas d'hier. Naturellement, je m'associe aux élus, qui sont aux élus, qui sont démunis, ainsi qu'aux habitants de Mayotte, pour demander au Gouvernement de rétablir l'ordre le plus rapidement possible. Vous revenez d'un déplacement important avec le ministre de l'intérieur et des outre-mer et nous sommes sensibles et attentifs aux annonces qui ont été faites. N'oublions pas que d'autres collectivités sont concernées par ces questions sécuritaires ou d'immigration incontrôlée. En Guyane et aux Antilles, l'État doit y apporter une réponse efficace pour protéger nos concitoyens et préserver l'attractivité de ces territoires. J'en viens maintenant à la vie chère, qui ne fait que s'accentuer dans nos territoires. Dans les outre-mer, la situation socio-économique est beaucoup plus fragilisée que dans le reste de la France. Lors de la rencontre organisée avec les maires ultramarins au Sénat, le 21 novembre dernier, de nombreux élus ont de nouveau sonné l'alerte quant à la dégradation du cadre de vie. de vie. Les plus modestes souffrent et sont les premiers touchés par ce fléau de la vie chère, amplifié, ces derniers mois, par la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières. Par ailleurs, il est inadmissible que nous n'ayons pas partout sur nos territoires accès à l'eau, aux soins ou encore à un logement décent- nous y reviendrons lors de l'examen des amendements. Enfin, comment ignorer le désarroi de nos compatriotes ultramarins face à l'explosion des prix des billets d'avion ? Notre délégation va se pencher

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d'entamer l'examen des crédits de la mission « Outre-mer », je tenais à saluer le fait que le Gouvernement ait abondé le budget initial d'un peu plus de 53 millions d'euros de crédits nouveaux, issus des amendements discutés en première lecture à l'Assemblée nationale. Cela va permettre de renforcer les moyens consacrés au dispositif Corom à l'attention des communes en difficulté, de consolider le développement du RSMA, de compenser la hausse du gazole pour les industries ultramarines, mais aussi d'améliorer les moyens alloués à la continuité territoriale. À périmètre constant, ce budget est donc en hausse d'un peu plus de 11

à des risques pour leur sécurité ou leur santé et entravent leur quotidien. De tels logements sont de plus en plus présents sur nos territoires. C'est la raison pour laquelle je propose, avec plusieurs de mes collègues, d'augmenter les crédits alloués à la résorption de l'habitat indigne et insalubre en outre-mer, qui ont été surconsommés l'an dernier.

nous devons assouplir les procédures, qui sont longues et complexes, et mettre en adéquation les financements avec les besoins réels. À La Réunion, par exemple, les Tl et les T2 sont construits en nombre insuffisant.

Pourquoi ne pas réfléchir à un bouclier qualité-prix sur les matériaux pour l'habitat ? Il est temps de redresser la barre afin de proposer aux Ultramarins une politique du logement ambitieuse et efficace.

des surcoûts. Ainsi, la ville de Saint-Pierre a contractualisé avec l'Anru en mars 2020, soit à la veille de la crise du covid-19. La ville se voit désormais contrainte de solliciter une modification du calendrier

Le logement, c'est, enfin, l'habitat individuel et collectif de nos seniors, qu'il faut adapter et rénover en innovant, pour le conformer à nos habitudes de vie.

portée sur les facteurs d'augmentation des prix. La quasi-totalité des élus ultramarins s'entend pour considérer que la remise en cause de l'octroi de mer constitue un danger grave pour les finances des collectivités locales, dans la mesure où les recettes de cette taxe peuvent représenter jusqu'à 40 % des budgets de fonctionnement des communes.

amenderont ces crédits alloués à l'outre-mer ; je forme le voeu que, si le Gouvernement devait de nouveau engager sa responsabilité sur la première et la seconde partie du PLF lors de la navette, certains des apports de la Haute Assemblée soient conservés. Tous nos

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette discussion budgétaire relative à l'outre-mer s'inscrit dans un contexte inflationniste et de renchérissement du coût de l'énergie, alors que nos concitoyens ultramarins sont déjà fragilisés par de nombreux facteurs : une balance commerciale déficitaire, des taux de chômage deux à trois fois plus élevés qu'en métropole ou encore un éloignement géographique favorisant la vie chère. Aussi, dans ce contexte particulier, les crédits de la mission « Outre-mer » doivent être mobilisés plus que jamais au service de nos territoires ultramarins. Il s'agit de donner à ces territoires les moyens de leur développement de les aider à relever les multiples défis auxquels ils sont confrontés. C'est donc avec satisfaction que je constate que ces crédits sont en légère augmentation par rapport à l'année 2022.

Toutefois, il faut souligner que la mission « Outre-mer » ne constitue qu'une petite partie du budget de l'État consacré aux territoires ultramarins. En effet, la politique transversale de l'État en direction de l'outre-mer est portée par 101 programmes relevant de 32 missions. L'effort budgétaire de l'État en faveur des territoires ultramarins s'élève ainsi à 20,1 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à 21,7 milliards d'euros en crédits de paiement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023. la hausse est-elle respectivement de 1,1 % et de 3,7 % par rapport à l'année 2022 ; elle est bienvenue, car les besoins sont importants. À cet égard, je tiens à évoquer la nécessité de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes Ultramarins. Depuis plusieurs années déjà, leur situation du point de vue de l'emploi suscite des inquiétudes ; elle doit être rapidement améliorée si l'on veut que soit garanti non seulement leur avenir, mais également le développement des outre-mer. Aussi, je me félicite de la hausse des crédits en matière de soutien à l'insertion et à la formation des jeunes Ultramarins- elle est de près de 10 % en autorisations d'engagement et de 13 % en crédits de paiement. Je veux également mettre l'accent sur l'état du parc de logements en outre-mer. Cette question est une préoccupation forte des Ultramarins et la situation de l'habitat indigne et insalubre impose une politique particulièrement volontariste. Aussi, je salue l'initiative de nos rapporteurs de majorer de 4 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement les crédits destinés à la résorption de l'habitat insalubre. Avant de conclure, je tiens à souligner un problème récurrent : la sous-consommation des crédits outre-mer. Cette situation est extrêmement dommageable eu égard aux besoins impérieux des territoires ultramarins, notamment en matière de logement et d'emploi. Il est primordial de trouver les moyens pour y remédier. Monsieur le ministre, mes chers collègues, les outre-mer, ce sont douze territoires français répartis sur les deux hémisphères et rayonnant sur trois océans territoires qui sont la France. Nous avons le devoir d'instaurer une égalité réelle entre tous nos territoires afin que chaque citoyen puisse y vivre avec le sentiment d'appartenir à une seule et même communauté. Ce budget y contribue. Aussi le groupe Les Indépendants votera-t-il les crédits de la mission « Outre-mer » du projet de loi de finances pour 2023. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission « Outre-mer » n'ont augmenté que de 1,71 % en autorisations d'engagement et de 1,29 % en crédits de paiement par rapport à la loi de finances pour C'est peu pour une mission dont le principal objectif est le rattrapage des écarts persistants entre l'outre-mer et la métropole, dans un contexte de crise économique et sociale, et alors que les inégalités entre les territoires ultramarins et la métropole ne cessent de se creuser.

Comme l'a montré le rapport que j'ai commis avec mes collègues Victorin Lurel et Micheline Jacques, que je salue, l'objectif de 10 000 logements créés ou réhabilités chaque année n'est, hélas ! pas atteint. Pourtant, 80 % des habitants des outre-mer sont éligibles au logement social ; mais seuls 15 % d'entre À cet égard, nous regrettons que les fonds demeurent insuffisants pour résorber l'habitat insalubre et que les crédits de l'action Logement du programme 123 baissent de 10,57 % en crédits de paiement. Plutôt que de lutter contre les facteurs de la sous-consommation des crédits outre-mer, on réduit les lignes budgétaires. Si les collectivités ultramarines ont leur part de responsabilité dans cette situation, le manque d'ingénierie de l'État et la faiblesse du pilotage du ministère sont également en cause, comme nous le soulignions dans notre rapport. Nous y demandions l'organisation d'assises du logement outre-mer ; monsieur le ministre, nous n'attendons que votre signal. Rappelons aussi que la Cour des comptes estimait, en septembre 2020, que les coûts des matériaux étaient de 20 % à 30 % supérieurs en outre-mer. Depuis lors, cet écart n'a fait que s'aggraver ; raison raison de plus, comme nous le suggérions également, pour renforcer les filières locales et pour promouvoir les matériaux biosourcés locaux et une architecture bioclimatique s'appuyant sur les savoir-faire traditionnels et l'habitat vernaculaire. Voilà une impulsion à donner pour utiliser les nombreux crédits non consommés d'un plan de relance ! Ce programme budgétaire a pour vocation d'opérer un rattrapage de niveau de vie ; et pourtant, il ne comprend toujours pas de plan Marshall des infrastructures,

Comment imaginer, dans la septième puissance économique mondiale, que des robinets soient à sec ou déversent une eau blanche saumâtre, voire contaminée au chlordécone ; que les coupures d'eau soient hebdomadaires, comme en Guadeloupe ; que des écoles ferment plus d'un mois par an faute d'eau ?

Cette catastrophe sociale se double naturellement d'une catastrophe écologique : le débit des rivières diminue dangereusement, ce qui menace la continuité écologique et des pans entiers de la biodiversité. Les nappes phréatiques, souvent contaminées au chlordécone, risquent en outre la salinisation.

Financement, ingénierie, main-d'oeuvre : l'État doit suppléer les collectivités locales partout où c'est nécessaire. Il faut mettre en place une gestion publique de l'eau et cesser de confier ce précieux commun à la prédation de Veolia et consorts. Un mot, pour finir, de la protection de la biodiversité ultramarine, qui concentre plus de 90 % des espèces présentes sur le territoire national. Selon les estimations de l'Office national de la biodiversité (OFB), ce sont 500 000 à 1 million d'espèces qui sont menacées de disparition. Monsieur le ministre, la visibilité fait grandement défaut, dans ce PLF, quant aux crédits destinés spécifiquement à la protection de la biodiversité ultramarine. Cela est d'autant plus problématique que la France vient d'annoncer un renforcement de ses aires marines protégées. En tout état de cause, ne serait-il pas préférable que la protection de la biodiversité ultramarine fasse l'objet d'un programme spécifique de la mission « Outre-mer » ? Avec toutes les réserves énoncées, et en souhaitant que les avancées du Sénat résistent au 49.3,

l'examen des crédits de la mission « Outre-mer » du projet de loi de finances est un moment toujours particulier pour nous, sénateurs ultramarins. Je dis « nous », parce que ces débats, s'ils sont scrutés dans nos territoires, n'attirent généralement pas les foules dans cet hémicycle. Les attentes et les enjeux sont pourtant nombreux, puisqu'il s'agit de combler le retard de développement pris sur l'Hexagone en matière d'emploi et de conditions de vie. Cette année, l'examen de la mission revêt peut-être une dimension supplémentaire. C'est en effet une année de renouvellement sénatorial, mais c'est aussi la première fois depuis deux ans que nous nous réunissons pour de ces crédits. Avec 2,75 milliards d'euros en autorisations d'engagement, le budget du ministère des outre-mer enregistre pour 2023 une légère hausse, de 1,7 %, par rapport à la loi de finances initiale pour 2022.

La hausse des crédits du programme 138 au titre de la compensation des exonérations de cotisations sociales patronales est bien sûr un motif de satisfaction elle permettra de renforcer la compétitivité des entreprises ultramarines et de soutenir l'emploi dans les secteurs stratégiques. Autre motif de réjouissance, la forte progression des moyens alloués à l'aide à l'insertion et à la qualification professionnelle, portée par le déploiement du plan SMA 2025+. Les quelque 30 millions d'euros supplémentaires qui seront mobilisés permettront de poursuivre les projets entrepris cette année, notamment à Mayotte et en Polynésie française. Ladom continuera de mettre en oeuvre l'accord-cadre national avec Pôle emploi et recentrera ses actions de formation sur des filières stratégiques et d'avenir comme la transition écologique et le numérique. Second volet de la mission, le programme 123, « Conditions de vie outre-mer », enregistre pour 2023 une hausse de 4 millions d'euros de la ligne budgétaire unique consacrée au logement social. Cette augmentation s'inscrit dans la dynamique impulsée par le plan Logement outre-mer 2019-2022, ce dont nous nous réjouissons. Ce budget

et le financement de la subvention à la collectivité territoriale de Guyane. Ce soutien aux collectivités se traduira également par un effort exceptionnel de 30 millions d'euros pour soutenir le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, je me félicite- j'y reviendrai dans quelques instants. Notons également la poursuite de l'action de l'État en matière d'assistance technique et de soutien à l'ingénierie pour la concrétisation des projets structurants des territoires ultramarins, ainsi que l'effort déployé pour répondre au au problème de la sous-consommation des crédits que nous votons chaque année. Au-delà de nos talents locaux, nos collectivités doivent se saisir des outils dont elles disposent- je pense notamment à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je me réjouis par ailleurs de la contribution du ministère à la lutte contre les algues sargasses et au programme d'intervention territoriale de l'État, ainsi que de la prise en charge de la totalité des investissements des services publics antisargasses qui viennent d'être créés en Guadeloupe et en Martinique.

mais aussi d'un engagement pluriannuel de l'État. C'est à mes yeux le seul moyen de retrouver la sérénité nécessaire et de régler définitivement cette question qui embrase un

En 2023, plus de 20 milliards d'euros seront ainsi mobilisés pour les outre-mer, en hausse de 1,1 % en autorisations d'engagement et de 3,7 % en crédits de paiement. C'est beaucoup, et pourtant, nous ne disposons pas, à ce jour, d'un espace de discussion sur ce budget transversal qui fonde le développement de nos territoires.

pouvoir un jour discuter de la réalité de nos territoires, de nos aspirations, de nos différences. En effet, les questions relatives à la sécurité, à l'éducation et à la santé, par exemple, ne se posent pas dans les mêmes termes que l'on soit à Mayotte, en Polynésie française ou en Guadeloupe.

La prise en compte de nos cultures, de nos expressions, de nos passés douloureux doit présider au traitement de notre quotidien. Votre budget est en augmentation, monsieur le ministre. J'aurais pu m'en contenter, m'en satisfaire ; mais non ! j'aimerais que l'on aille plus loin.

je vous demande notamment de sanctuariser une somme pour l'accompagnement dans le logement social. Les bailleurs sociaux sont aux abois, non parce qu'ils n'auraient pas assez de sous pour construire, mais parce qu'ils sont désormais confrontés à l'immense difficulté du vivre-ensemble.

85 % d'entre eux veulent rentrer dans leur pays. Nos peuples ont soif d'entendre des mots forts, des intentions fermes, des objectifs évaluables

Ne sanctionnez pas systématiquement nos propositions pour un droit au bonheur de nos compatriotes d'un implacable et froid avis défavorable

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à souligner l'augmentation de plus de 2,7 milliards d'euros en autorisations d'engagement des crédits alloués à la mission « Outre-mer ». Les dispositifs de soutien exceptionnel aux collectivités d'outre-mer sont renforcés, ce qui permet d'élargir la liste des bénéficiaires. Cela témoigne de la bonne volonté du Gouvernement de se soucier- enfin -de tous les territoires de la République. Mais est-ce suffisant pour faire face à l'ampleur des enjeux et de la détresse, évoquée à l'instant, des habitants des outre-mer ? La première journée du 104 Congrès des maires, à Paris, était consacrée à l'outre-mer.

Dans ces territoires doublement affectés par la crise économique, énergétique, écologique, sanitaire, et dont le retard de développement ne pourra pas être compensé de sitôt, les communes et les élus locaux ont besoin d'un accompagnement fort pour mettre en place des politiques publiques, pour exercer leur mission première de service public et pour lutter contre la pauvreté grandissante. L'inflation a dépassé les 10 %. La vie est chère, le pouvoir d'achat diminue, la population est en détresse. Les mobilisations populaires continuent, et le calme n'est malheureusement pas près de revenir. Les produits alimentaires sont entre 28 % et 38 % plus chers qu'en métropole. Le taux de pauvreté en outre-mer varie entre 33 % et 77 %, contre 14 % dans l'Hexagone. Les citoyennes et les citoyens des outre-mer demandent une égalité de traitement et veulent qu'on les considère comme tous les autres. Pour cela, ils et elles doivent pouvoir travailler et vivre dignement ; l'emploi est un vecteur fondamental de lutte contre cette pauvreté. Mais le niveau

L'égalité républicaine doit exister pour toutes et pour tous. Ces territoires veulent se développer, avoir leur destin en main. Les jeunes veulent étudier dans de bonnes conditions, s'insérer dans le milieu professionnel, dépasser ce plafond de verre et construire leur vie. Ils ont besoin de soutien et d'écoute. Monsieur le ministre, ce ne sont pas des décisions prises d'« en haut » qui permettront de comprendre les problématiques du « bas ». Il faut faire avec celles et ceux qui sont confrontés aux difficultés quotidiennes. Il faut faire avec les maires, avec les élus dans leur diversité, qui demandent un dialogue et de la coopération. Les représentants de l'État doivent entendre les revendications et adapter leurs propositions en fonction des territoires.

à peine du Caillou, où avec M. Darmanin, ministre de l'intérieur et des outre-mer, il a travaillé au retour du dialogue entre tous les partis calédoniens, indépendantistes et non indépendantistes. C'est très important à ce moment de notre histoire Votre présence témoigne de votre considération pour la représentation sénatoriale. Le projet de loi de finances que nous examinons traduit l'intention du Gouvernement d'aider nos compatriotes ultramarins à faire face à un contexte international particulièrement défavorable, qui aggrave les difficultés déjà considérables de nos territoires. Je salue en particulier les moyens alloués au plan SMA 2025+ ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique dans le Pacifique. Monsieur le ministre, mon propos sera précis : il faut désormais traduire dans les faits l'une des recommandations du rapport d'information de l'Assemblée nationale en date du 3 octobre 2019 sur la continuité territoriale dans les outre-mer. J'invite donc le Gouvernement à appliquer effectivement l'article L. 1803-4 du code des transports sur l'aide à la continuité territoriale. À l'heure

pour la Polynésie française, dont le territoire intérieur est composé de 118 îles réparties sur 5,5 millions de kilomètres carrés. cela vaut, bien sûr, pour les îles de l'archipel calédonien, les populations de Lifou, de Maré, de Tiga, d'Ouvéa, de Bélep

ont impérativement besoin de rejoindre régulièrement l'île de Wallis, distante de 250 kilomètres. Et certains services, notamment médicaux, ne sont accessibles aux habitants de Wallis de Futuna que s'ils se rendent à Nouméa, distante de 2 100 kilomètres. L'extension de l'aide à la continuité territoriale aux déplacements inter-îles permettrait d'éviter l'exode des populations vers Papeete et Nouméa et d'assurer le développement économique et le désenclavement de ces territoires.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen des crédits de la mission « Outre-mer » est l'occasion pour moi de vous livrer l'état d'esprit de nombreux collègues des territoires ultramarins. Si nous pouvons nous féliciter d'un budget en augmentation et du soutien d'un ministre qui connaît et apprécie nos territoires,

Comment expliquer que les gens continuent à mourir à Saint-Martin faute de pouvoir être transférés vers le CHU le plus proche après dix-huit heures ? Une solution n'a toujours pas été trouvée pour garantir ces évacuations sanitaires, par exemple en autorisant les vols après dix-huit heures au départ de l'aéroport de Grand-Case.

conformément aux recommandations de la mission interministérielle de juillet 2015, mais aussi au référé de la Cour des comptes en date du 22 décembre 2017. enfin, le réengagement de l'État dans l'administration des douanes. Il ne reste que deux douaniers à Saint-Martin, monsieur le ministre ! Cela signifie qu'il n'y a plus de contrôle effectif sur le territoire. Saint-Martin a été érigée en collectivité d'outre-mer au sens de l'article 74 de la Constitution, notre statut, au sens du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'a pas été modifié.

Ne laissez pas la géographie décider de qui est citoyen français à part entière, ou entièrement à part ! Très bien

Monsieur le ministre, le budget est en augmentation. Sera-t-il à la hauteur des besoins et des enjeux qui s'imposent aux élus ultramarins ? Telle est la question. Je souhaite insister sur certaines problématiques qui sont malheureusement toujours d'actualité et qui me tiennent particulièrement à coeur.

: lors du dernier congrès des maires, ils ont mis en évidence les problématiques qui leur sont propres. Aussi, monsieur le ministre, il serait souhaitable que le Gouvernement prenne en compte ces différents éléments en fonction des besoins spécifiques de chacun de nos territoires, pour que nous puissions tous ensemble bénéficier de son accompagnement. La parole

C'est déjà beaucoup d'être derrière et je ne tiens pas à être devant. La première priorité, c'est de répondre aux préoccupations du quotidien, en accordant une attention particulière aux sujets environnementaux.

création de valeur dans chaque territoire. Les contrats de plan arrivent à échéance en 2022. Ils seront prolongés par avenant en 2023, avec une contribution stabilisée de l'État. C'est tout de même un effort budgétaire de 530 millions

je veux insister sur la prolongation de la défiscalisation jusqu'en 2029, qui a été décidée pour tous les dispositifs et tous les territoires : c'est un geste fort que vous avez été nombreux à demander pour donner de la visibilité aux investisseurs.

Les moyens de mon ministère qui y sont dédiés passeront de 205 à 270 millions d'euros en 2023, soit une de 32 % : le maire de mon village de Langogne n'en revient pas ! Certes, il y a du retard à rattraper, mais enfin, Langogne, ce n'est pas non plus Abou Dhabi ! C'est une progression considérable que nous avons fortement défendue avec Gérald Darmanin

d'outre-mer (Dacom), conformément à l'engagement du Président de la République : depuis 2016, ce rattrapage s'élève à 150 millions d'euros. Les collectivités ultramarines profiteront aussi de la progression nationale de la dotation globale de fonctionnement,

et de mettre en place des prérequis pour une planification pluriannuelle afin de mieux répondre aux besoins des collectivités et de nos concitoyens des outre-mer, en toute transparence. L'amendement n° II-809

millions d'euros les crédits du programme 123, « Conditions de vie outre-mer », pour accroître les moyens dédiés à la continuité territoriale. Pour l'année 2022, Ladom estime estime l'augmentation du prix des billets d'avion à environ 23 %, ce qui l'a conduite à puiser dans sa trésorerie. Dans ce contexte, il paraît indispensable de donner les moyens à Ladom de remplir effectivement ses missions, qui relèvent de l'unité de la République et de la solidarité vis-à-vis des citoyens ultramarins. Cet amendement vise tout particulièrement à interpeller le ministre chargé des outre-mer pour qu'il confirme l'engagement pris à l'Assemblée nationale et qu'il en tire les conséquences en actualisant au plus vite l'arrêté du 18 novembre 2010 fixant les montants des différentes aides à la continuité territoriale. Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement tend à prélever 1 million d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le programme 138 pour abonder le programme 123 de la mission « Outre-mer ». L'amendement : La parole est à Mme Annick Petrus. Cet amendement a pour objet d'abonder de 350 000 euros les crédits consacrés à la continuité territoriale, afin de permettre une prise en charge des frais de transport et des indemnités forfaitaires journalières d'hébergement des malades résidant sur le territoire de Saint-Martin et devant se rendre en Guadeloupe, en Martinique, ou encore plus loin, dans l'Hexagone pour y être soignés, faute de structures ou de spécialistes sur le territoire. Il me paraît nécessaire de rappeler l'importance du volet santé de l'aide à la continuité territoriale. Au sein du budget de la mission « Outre-mer » pour 2023, les crédits consacrés à la continuité territoriale ne permettent pas de prendre en charge ces frais, pourtant élevés pour les Ultramarins : ils doivent les financer à partir de leur budget personnel afin d'éviter une rupture ou une perte de chance dans leur parcours de soin. En effet, sur le territoire le territoire de Saint-Martin, nous n'avons pas de service de chirurgie vasculaire, ni de chirurgie plastique de reconstruction, ni de neurochirurgie, ni de chirurgie cardiaque. Au niveau des spécialités médicales, il manque un spécialiste en neurologie ou en rhumatologie ; nous ne comptons ni pneumologue ni chirurgien spécialisé de l'épaule, et Autant de médecins qui ne sont pas présents ou qui ne viennent plus, pour ceux qui faisaient le déplacement, car le coût du billet d'avion, en constante augmentation, les en aura définitivement dissuadés. Il en est de même pour les patients qui ne peuvent se rendre en Martinique, en Guadeloupe, ou en France hexagonale en raison du coût du transport. Le fonds de de continuité territoriale doit donc pouvoir prendre en charge, sans condition de ressources, les titres de transport pour ces déplacements entre les collectivités de résidence outre-mer et l'Hexagone, lorsque la santé du patient le nécessite.

ou à une autre structure ? Cette question doit également être posée. Par ailleurs, d'après nos informations, la délégation sénatoriale aux outre-mer devrait conduire une mission d'information sur la continuité territoriale, dès l'année prochaine. Il nous paraît raisonnable d'attendre ses conclusions et ses recommandations.

les crédits alloués à la continuité territoriale étaient majorés de 5 millions d'euros, afin de réellement garantir le principe de continuité territoriale, dans un contexte inflationniste- que vous avez évoqué -caractérisé par une hausse des prix des billets d'avion pour les trajets entre la métropole et les territoires d'outre-mer, hausse d'environ 20 % en un an. % en un an. Cette augmentation de plus de 10 % des crédits dédiés à la continuité territoriale semble déjà de nature à répondre aux hausses attendues des prix des billets d'avion. De surcroît, contrairement à d'autres actions, les crédits de l'action n° 03 du programme 123 sont, de manière régulière, sous-consommés. Je ne fais pas référence aux années 2020 et 2021 marquées par la crise sanitaire, qui ont, de fait, vu le nombre de vols entre la métropole et les outre-mer diminuer fortement.

2022, concerne non pas les billets d'avion, mais la desserte maritime exercée dans le cadre de la délégation de service public. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes sujets. Nous restons vigilants, comme vous, à la hausse des prix des billets d'avion et à la consommation des crédits dédiés à la continuité territoriale. Nous n'hésiterons donc pas à demander une majoration en 2024,

rectifié de Mme Petrus vise à majorer de 350 000 euros les crédits du programme 123, afin de financer la prise en charge du transport et des indemnités forfaitaires journalières d'hébergement des personnes malades

d'avion. Le baromètre du transport aérien nous indique que, au départ de l'ensemble des départements d'outre-mer, l'augmentation des prix des billets d'avion atteignait 32,4 % au mois d'octobre 2022, et 19,2 % au cumul. Cette tendance touche les quatre départements de manière différenciée, la Guadeloupe- que je connais mieux -affichant la plus forte progression, soit 37,2 %.

de vote. Je vais peut-être décevoir M. le ministre, mais l'article L. 1803-1 du code des transports prévoit que la politique de continuité territoriale « tend à atténuer les contraintes de l'insularité et de l'éloignement et à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé

L'accompagnement des malades est assuré par la sécurité sociale, qui prend en charge le prix du billet d'avion du malade et celui d'un accompagnant, ou encore

dans la perspective d'un règlement global de ce sujet.

de l'instabilité politique, il était impératif de réformer ces régimes pour les adapter aux nouvelles exigences économiques, démographiques et de santé publique. La population de Polynésie française est de plus en plus vieillissante et touchée par de graves pathologies, dont le coût de gestion est extrêmement onéreux pour cette petite collectivité. Les petite collectivité. Les charges liées aux maladies radio-induites, résultant des essais nucléaires, des ressortissants de la CPS obèrent gravement le régime maladie de la caisse. L'impact financier a été évalué à plus de 47 millions d'euros

de l'État de 2015 à 2020, dans le cadre d'une convention solidarité signée entre l'État et le pays. Depuis lors, des réformes essentielles ont été engagées localement pour une meilleure gouvernance de la CPS et par la mise en place d'une nouvelle TVA sociale afin d'assurer l'équilibre financier des différents régimes de prestations sociales.

enveloppe a permis d'améliorer la situation de neuf communes contractantes- Sada à Mayotte, Saint-Benoît à La Réunion, Cayenne et Iracoubo en Guyane, Pointe-à-Pitre, Saint-François et Basse-Terre en Guadeloupe, ainsi que Fort-de-France et Saint-Pierre à la Martinique

Pourtant, dans l'ensemble des Drom, l'encours de dette a augmenté de 36,6 % entre 2016 et 2021, passant de 2 376,2 à 3 246,5 millions d'euros. sur la période 2016-2022, les ressources d'investissement ont baissé de 31,47 % pour des charges d'investissement restées stables. Cette situation a pour conséquence l'allongement des délais de paiement.

Merci

Il est certain qu'une stratégie générale pourrait favoriser le retour des jeunes Ultramarins partis, notamment pour étudier, en métropole ou à l'étranger. Mais ce qui fera avant tout revenir les jeunes actifs, ce sont des logements abordables, des débouchés professionnels et un accès aux services publics équivalent à celui autant d'actions qui sont l'objet même de la mission « Outre-mer ». Faut-il oeuvrer encore en ce sens ? Évidemment, oui : le rattrapage des niveaux et conditions de vie entre l'outre-mer et la métropole est un préalable nécessaire au retour des jeunes Ultramarins.

Cet amendement vise à majorer de 5 millions d'euros les crédits de la LBU afin de créer un volet social permettant d'accompagner les bailleurs sociaux. Je comprends parfaitement les préoccupations des signataires de cet amendement : il faut effectivement saluer le travail des bailleurs qui ont tenté, sur leurs fonds propres, de déployer des solutions. Toutefois, ces dernières ne peuvent qu'être provisoires et incomplètes.

engendré un accroissement des demandes de financement le dispositif de PDOM émises par les entreprises ultramarines, qui ont rencontré des difficultés financières. Il nous apparaît donc que la consommation de ces crédits est très sensible à la conjoncture économique. Or, dans le contexte économique actuel, la situation des entreprises devrait

Cet amendement vise à augmenter de 4 millions d'euros les crédits dédiés à la résorption de l'habitat indigne et insalubre en outre-mer. Les crédits alloués à cette action sont stables depuis plusieurs années, à hauteur de 20 millions d'euros en crédits de paiement Or les Drom présentent une proportion de logements indignes et insalubres nettement supérieure à la métropole : ils représenteraient près de 19,4 % du parc de logements, soit environ 150 000 habitations sur les 774 641 résidences principales que compte le parc, contre 1,2 % en France métropolitaine.

Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement

Par ailleurs, si cette problématique est prégnante à Mayotte, elle touche également de nombreux citoyens français, quel que soit leur lieu de résidence. Aussi, la réponse doit être globale, au même titre que les aides apportées aux ménages face à la hausse des prix de l'énergie.

Les violences intrafamiliales sont un sujet sensible, qui doit tous nous mobiliser. En outre-mer, selon l'Insee, ces violences, mesurées à partir des dépôts de plainte, sont encore plus répandues que dans l'Hexagone.

Il faut lutter contre ce phénomène, c'est une évidence. Pour autant, je ne pense pas que les crédits de la mission « Outre-mer » soient le meilleur vecteur pour renforcer cette lutte. Actuellement, les crédits alloués aux actions de lutte contre les violences intrafamiliales sont portés par les services de

À Mayotte, par exemple, chaque année, environ 650 femmes franchissent courageusement la porte du commissariat de Mamoudzou ou d'une brigade de gendarmerie de l'île pour signaler des violences conjugales. Seuls 150 de ces signalements donnent lieu à des procédures judiciaires. Des moyens sont mis en oeuvre pour aider les victimes et sensibiliser les professionnels aux spécificités

joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en outre-mer comme en métropole. Néanmoins, les efforts doivent se poursuivre et les moyens être renforcés afin de lutter contre les violences intrafamiliales en outre-mer, pour que l'accueil, l'orientation et la protection des victimes soient plus efficaces.

des victimes. Monsieur le ministre, je crois savoir qu'un texte est en cours de préparation avec la ministre Isabelle Rome. Je vous adresse à ce sujet une demande formelle et appuyée : associez les parlementaires ultramarins à son élaboration, pour prendre en compte nos spécificités.

Par ailleurs, Saint-Pierre-et-Miquelon a également signé un contrat de convergence et de transformation, pour un montant de 9,5 millions d'euros, qui a permis, entre autres choses, de financer des études et aménagements pour le barrage de la Vigie, la route de l'isthme à Miquelon et la route littorale de Saint-Pierre. La renégociation de ce contrat, prévue en 2023, pourrait être l'occasion de prévoir les crédits pour les travaux nécessaires à la protection du littoral, mais les crédits ne seraient alors disponibles qu'en 2024. C'est pourquoi nous sollicitons l'avis du Gouvernement sur cet amendement. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Saint-Laurent-du-Maroni et son environnement, mais aussi les autres territoires, y compris maintenant de plus en plus la Guadeloupe. Quel est l'avis de la commission ? ? Le fonds de coopération régionale, qui est doté d'un peu moins de 1,5 million d'euros par an, vise essentiellement à mettre en place des actions de coopération économique, sociale et culturelle avec les autres pays des régions ultramarines. À ce jour, il n'a pas de compétence

Ainsi, les crédits existent et nous avons formulé des recommandations pour qu'ils soient pleinement consommés. Soyez assurés que nous y serons attentifs. Quand le FEI sera intégralement consommé chaque année, nous pourrons légitimement demander une augmentation des crédits ouverts à ce titre, notamment pour des investissements liés à l'accès à l'eau potable.

Il s'agit de demander un meilleur investissement de l'État au sein des départements d'outre-mer, notamment en Polynésie française. Le fonds intercommunal de péréquation (FIP) ayant diminué, le service de public de l'eau est remis en cause. Les communes n'ont pas les moyens nécessaires pour assurer la maintenance des réseaux d'adduction d'eau, qui est une compétence communale.

à régler ce sujet majeur pour la Polynésie française, vous faites une erreur. Permettez-moi de vous le dire en tant qu'élu de la Polynésie française et de la République.

En effet, pour qu'un rapport soit utile, il faut qu'il soit complet et instruit dans de bonnes conditions. Dans ce contexte, le délai de trois mois proposé paraît court ; il est donc proposé de le porter à six mois.

même s'il n'est pas en lui-même parfait- la perfection est-elle de ce monde ? -, ce budget a le mérite de répondre partiellement à des questions pour lesquelles nous avons le même intérêt et sur lesquelles nous portons un diagnostic commun.

-et poser un regard plus objectif sur la qualité du travail que produit notre enseignement scolaire. Les résultats ne sont pas tragiques, ils ne sont pas à la hauteur des ambitions d'un grand pays comme le nôtre, particulièrement dans le domaine des sciences et des mathématiques. Monsieur le ministre, je

et de rappeler aux chefs d'établissement qu'ils seraient évalués. Dans les faits, le rythme est beaucoup plus lent, puisque seulement 5 % des établissements ont été évalués.

Parce que vous poursuivez cet effort et acceptez l'idée que l'enseignement français, aussi superbe et fort de ses traditions et de son histoire

avons donc le devoir absolu de nous poser la question du statut de l'enseignant. De ce point de vue, les comparaisons internationales qu'a lancées la commission des finances sont assez cruelles pour notre conservatisme tranquille et heureux, mais décalé des réalités.

les conséquences pratiques d'une tragédie française, à savoir son échec démographique. Le débat qui s'amorce nous permettra d'en parler entre nous, en particulier avec la majorité sénatoriale que je voudrais convaincre

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, les crédits de la mission « Enseignement scolaire » s'établiront en 2023 à plus de 58 milliards d'euros, soit une hausse de 3,5 milliards d'euros.

Enseignement agricole », doté pour 2023 de 1,59 milliard d'euros, soit une augmentation de 67,8 millions d'euros par rapport à 2022. Au-delà de la hausse attendue des dépenses de personnel, qui découle notamment de la revalorisation du point d'indice, l'augmentation des crédits de la mission se caractérise surtout par un bel effort en faveur de l'école inclusive, à hauteur de 10,28 millions d'euros supplémentaires pour 2023, le nombre de jeunes en situation de handicap accueillis dans l'enseignement agricole ayant encore progressé de 26 % cette année.

Je tiens cependant à vous alerter sur les chiffres de la rentrée 2022. Le nombre d'élèves scolarisés au sein des établissements de l'enseignement technique agricole est en baisse de 1,1 % cette année, soit une diminution de 1 743 élèves. La situation des brevets de technicien supérieur agricole (BTSA) est particulièrement inquiétante, puisque les effectifs dans ces formations, qui ont pourtant fait leurs preuves, ont diminué de 12,8 par rapport à la rentrée précédente. Il me semble indispensable de mettre en place au plus vite un groupe de travail afin de revaloriser le BTSA et de lui redonner une perspective claire, dans une dynamique bac+3.

Il est indispensable de mieux cerner les attentes des jeunes et d'encourager les établissements à se saisir, à leur échelle, de ces enjeux, en y associant leurs élèves. L'enseignement agricole se distingue encore cette année par l'excellence de ses résultats. Ses taux d'insertion professionnelle sont très élevés et son caractère innovant est reconnu. Cette qualité d'enseignement doit faut s'en inspirer, monsieur le ministre de l'éducation nationale ! Enfin, je terminerai en attirant votre attention sur la nécessité, plus que jamais, d'accompagner les établissements de l'enseignement technique agricole face à un contexte énergétique tendu et à une hausse globale des coûts de production, notamment alimentaires. Les établissements de l'enseignement technique agricole sont particulièrement énergivores, énergivores, en raison du fort taux d'élèves en internat : 57 % des élèves de l'enseignement technique agricole sont internes, souvent même le week-end. Il me semble donc essentiel de soutenir au plus vite les établissements de l'enseignement technique agricole, publics et privés, afin de leur permettre d'absorber les retombées de l'inflation, qui mettent gravement en péril leur trésorerie pour les mois à venir. Il existe déjà une solution simple pour les maisons familiales et rurales et les établissements privés agricoles du temps plein : il ne faut pas leur demander le remboursement des subventions de fonctionnement non consommées cette année loi de finances pour 2022. Néanmoins, en raison d'une augmentation satisfaisante du budget consacré à l'enseignement technique agricole, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis, à la suite de mon rapport, un avis favorable sur l'adoption des crédits du programme 143 consacré à l'enseignement agricole. Mes chers

L'école, creuset républicain cristallisant la convergence des valeurs fondatrices de notre société- l'humanisme, l'universalisme et le progrès -se doit de refléter la maxime : « La fin justifie les moyens. Monsieur le ministre, je crois en la sincérité de votre engagement pour la revalorisation de l'enseignement, la réussite de tous les élèves et une école innovante et inclusive luttant contre toutes les inégalités. Vous prolongez la dynamique engagée depuis 2017 en augmentant de manière inédite les crédits de la mission, de l'ordre de 6,5 % par rapport à 2022. Néanmoins, je ferai quelques observations. de finances prévoit des crédits significatifs afin d'améliorer la rémunération des enseignants, le retard accumulé était considérable. Il est donc essentiel que ce choc d'attractivité se poursuive. Le métier d'enseignant traverse une crise sans précédent ; les difficultés de recrutement ne sont pas seulement d'ordre financier. Le manque de considération sociale et de soutien hiérarchique, ainsi que des conditions d'exercice dégradées dans certains territoires expliquent la désaffection Les chiffres ont été rappelés : en 2018, 135 000 candidats se présentaient encore aux concours de la fonction publique de l'éducation nationale. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 90 000. Plus grave encore, les postes n'ont été couverts qu'à 83 % en 2022 par les candidats ayant été admis. Le recours croissant aux contractuels présente un intérêt en ce qu'il permet de combler un manque et de réadapter progressivement les effectifs aux besoins réels. Cependant, n'est-il pas antinomique de pallier les pénuries d'enseignants en recrutant des contractuels dont les qualifications sont plus que variables, quand, parallèlement, la formation initiale se tourne vers des compétences professionnelles renforcées ? La revalorisation des rémunérations, qui constitue l'essentiel de la hausse des crédits de la mission, ne doit être que le premier pas vers un objectif plus large de reconnaissance économique et sociale du corps enseignant. Rappelons que, en 1990, un professeur des écoles débutant touchait 1,8 fois le Smic, contre 1,5 fois aujourd'hui. En fin de carrière, un agrégé de classe exceptionnelle touchait alors 4,6 fois le Smic, contre 3,3 fois actuellement. Notons également que la rémunération d'un professeur des écoles est inférieure au salaire moyen des fonctionnaires civils de catégorie B. La comparaison avec nos confrères européens est également inquiétante tant le fossé s'est creusé. Les enseignants français commencent et terminent leur carrière avec un salaire inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Dans le contexte inflationniste inédit que nous connaissons, cette revalorisation est souhaitable, mais, au-delà de la conjoncture, elle est bien évidemment une affaire de statut. Mon autre interrogation concerne les accompagnants des élèves en situation de handicap

Nous faisons face à une augmentation spectaculaire du nombre d'élèves en situation de handicap, qui sont au nombre de 430 000 aujourd'hui, soit deux fois plus qu'il y a dix ans. Dans ces conditions, la création de 4 000 postes d'AESH constitue un effort substantiel. Cependant, compte tenu des conditions de travail précaires et des faibles rémunérations, de nombreux postes ne sont actuellement pas pourvus. En Seine-Saint-Denis, ce sont ainsi 1 000 emplois qui n'avaient pas trouvé preneur à la rentrée 2022.

par ailleurs un problème de cohérence entre la politique des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les capacités de l'éducation nationale à accueillir et à gérer financièrement ce dispositif. Espérons que la création de ces postes supplémentaires sera non pas un simple effet d'affichage, mais le point de départ d'une meilleure coopération entre ceux qui prescrivent et ceux qui organisent, ainsi que d'une plus grande considération pour une profession aujourd'hui indispensable. Enfin, je reviendrai sur la volonté d'anticiper les grandes évolutions démographiques en cours, qui ont des répercussions sur le nombre d'élèves scolarisés en France. Si le taux d'encadrement s'améliore, la France se caractérise toujours par un nombre d'enfants par classe nettement supérieur à la moyenne européenne, particulièrement dans le premier degré. Dans le contexte tendu que je rappelais, où le nombre de postes à pourvoir n'est pas comblé par les lauréats des concours, le principe de réussite pour tous n'est que trop vacillant.

La France est également le pays d'Europe où il y a le plus de problèmes de discipline. Dans l'OCDE, seuls le Brésil et l'Argentine font pire. Les atteintes à la laïcité se multiplient.

comment vous entendez, au-delà du salaire, accompagner l'entrée dans le métier des enseignants, moment crucial et sensible de leur carrière ! Comment allez-vous mettre un terme au bizutage institutionnel des néo-titulaires, qui prennent leur premier poste dans les zones les plus difficiles, sans accompagnement spécifique ? ? Allez-vous créer des postes à profil et des contrats de mission pour que les carrières soient moins linéaires ? Allez-vous enfin prendre en considération les secondes carrières ?

vous voulez donner plus de liberté et d'autonomie aux établissements et à leurs enseignants, et vous avez raison ! Les établissements, les professeurs et les élèves ont besoin de confiance en leurs initiatives.

Peut-on favoriser l'autonomie sans remettre en cause l'armature rigide du collège unique et sans étendre l'expérimentation du dispositif des « 6 tremplin » ? Peut-on redresser notre école sans la recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la transmission des savoirs fondamentaux ? Peut-on réaffirmer sa mission première

Monsieur le ministre, certes, vous additionnez des volontés multiples pour répondre à des problèmes qui ont une résonance dans l'opinion. Mais est-ce là une politique à la hauteur des enjeux ?

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, le métier d'enseignant est souvent considéré comme le plus beau métier du monde. Marcel Pagnol décrivait malicieusement les professeurs oeuvrant « aux quatre coins des départements pour y lutter contre l'ignorance et glorifier la République Cette belle définition est toujours d'actualité. Pourtant, force est de constater que ce métier semble aujourd'hui être victime d'un désamour profond. Je suis particulièrement préoccupée par la crise du recrutement, très visible dans l'enseignement scolaire.

Les témoignages de directeurs d'établissements se sont accumulés au cours des derniers mois pour alerter sur le manque de personnel. Aujourd'hui, c'est la question des démissions qui remonte. Le recours aux contractuels ne représente pas une solution satisfaisante à long Les conditions de travail, les évolutions de carrière proposées, la mobilité géographique et la rémunération sont autant de sujets majeurs dont nous devons nous saisir. Pour y répondre, le présent projet de loi de finances consacre plus de 1,1 milliard d'euros à la hausse des rémunérations du personnel de l'éducation nationale. En outre, comme cela a été annoncé pendant la campagne présidentielle, 300 millions d'euros sont destinés aux enseignants qui acceptent d'effectuer des missions complémentaires. Je tiens à souligner cet effort. Il s'ajoute aux avancées permises par le Grenelle de l'éducation. ailleurs, environ 60 % des enseignants pourront bénéficier de la prime d'activité au cours de l'année 2023. Enfin, de nouvelles mesures de revalorisation salariale ont été annoncées pour les enseignants débutants à partir de la rentrée 2023.

C'est un effort considérable, que je salue. Les crédits destinés à l'école inclusive augmentent également. On parle de 2,4 milliards d'euros

des élèves en situation de handicap ne bénéficient pas d'un accompagnement dédié. Cela ne peut plus durer. Nous devons rendre ce métier plus attractif et améliorer les conditions de travail, car les AESH sont les chevilles ouvrières de l'école inclusive. Nous pouvons également nous satisfaire de l'accueil d'environ 20 000 jeunes Ukrainiens au sein de nos écoles. Les académies de Nice et de Versailles sont en première ligne. Les retours sont positifs et je salue l'implication du corps enseignant pour permettre à ces jeunes élèves de se sentir les bienvenus dans nos écoles.

Cette décision va dans le bon sens et doit s'accompagner de décisions fortes pour relever le niveau moyen des élèves. Enfin, je salue votre engagement, monsieur le ministre, dans la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Rappelons qu'un jeune sur dix est victime de harcèlement. Nous devons oeuvrer collectivement pour permettre à tous les établissements de protéger leurs élèves. C'était l'objet de notre échange lors de votre venue au collège Louis-Braille à Esbly, en Seine-et-Marne.

à partir du jeudi 10 novembre. La lutte contre ce phénomène doit faire partie de nos priorités dans les années à venir. J'y suis particulièrement attachée, car l'école doit préparer les élèves à vivre dans une société bienveillante, en respectant autrui.

Il faut naturellement se réjouir de cette hausse, mais celle-ci ne parvient malheureusement pas à masquer la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouve l'éducation nationale dans notre pays. Monsieur le ministre, vous avez hérité d'un ministère qui a beaucoup souffert du passage de votre prédécesseur, enfermé qu'il était dans ses conceptions archaïques de l'éducation, éloignées des difficultés de terrain. attendions donc une rupture. Concernant les enseignants, la situation atteint un seuil critique, car l'éducation nationale ne parvient plus à recruter.

Si le Président de la République a annoncé qu'aucun enseignant ne démarrerait sa carrière en dessous de 2 000 euros net, la revalorisation sera en partie conditionnée à l'accomplissement de nouvelles tâches. Nous proposerons d'aller beaucoup plus loin par voie d'amendement.

Pourtant, leur rémunération est indigne : elle s'élève en moyenne à 850 euros par mois, soit un montant très largement inférieur au seuil de pauvreté, qui se situe aux alentours de 1 000 euros. Comment l'État employeur peut-il être un tel moteur de souffrance et fabriquer des travailleurs pauvres ?

à tel point que certaines écoles acceptent désormais que les enfants dont les parents peuvent se le permettre aient recours à des prestataires privés au sein des écoles de la République. Cette rupture d'égalité inacceptable doit nous alerter. Monsieur le ministre, il faut tout revoir : le statut des AESH, leur rémunération, leur formation, leurs conditions de travail. Sur ce sujet également, nous vous proposerons des amendements. Vient ensuite la question de l'enseignement professionnel. Les moyens qui lui sont consacrés augmentent seulement de 5,3 % en 2023, soit moins que l'inflation. De plus, cette branche souffre d'un manque chronique de moyens. Elle n'a cessé d'être détricotée par les réformes successives : moins d'établissements, moins d'élèves, moins d'heures d'enseignements, moins d'enseignants. En 2023, cette dynamique ne s'arrêtera pas, puisque le Gouvernement prévoit de supprimer 480 postes supplémentaires dans le second degré. Cette année, l'enseignement professionnel a également droit à une double tutelle, puisqu'il est désormais également rattaché au ministère du travail. Ce choix politique traduit une volonté de répondre aux besoins immédiats des entreprises, une volonté de soumission des parcours des élèves au marché du travail. Or l'éducation nationale- que je sache, l'enseignement professionnel en fait toujours partie -, ce n'est pas la soumission, c'est au contraire l'émancipation l'éducation nationale est de donner aux élèves les moyens de s'épanouir, d'apprendre et de prendre en main leur avenir, dans la voie qu'ils ont eux-mêmes choisie. Là encore, notre vision est antinomique de la vôtre, monsieur le ministre. Pour l'enseignement technique agricole, ce projet de budget met enfin un terme à trois années successives de baisse des effectifs d'enseignants, mais cela ne suffit pas. Il faut rebâtir, recruter, revaloriser, octroyer de nouveaux moyens.

au travail de la terre ; c'est là aussi le rôle de l'éducation nationale. En conclusion, monsieur le ministre, nous avons accueilli avec soulagement la fin des années Blanquer, qui ont été une catastrophe pour l'éducation nationale. projet de budget devait incarner votre nouvelle ambition, un nouvel élan pour votre ministère, mais le compte n'y est manifestement pas.

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, pendant deux ans, la crise sanitaire a profondément bouleversé notre système scolaire. Si la rentrée 2022 a marqué un retour à la normale, c'est grâce à la mobilisation des services de l'éducation nationale et aux enseignants, dont je veux ici saluer l'engagement. Il n'en demeure pas moins que le métier d'enseignant souffre d'un manque d'attractivité, dont nous connaissons tous ici les symptômes. La baisse continue du

Sans aucun doute, le manque de reconnaissance sociale, l'isolement ou les difficultés rencontrées dans la formation initiale et continue y sont pour quelque chose. Mais ne nous voilons pas la face : la première cause de cette désaffection croissante est le niveau de rémunération des enseignants. ce projet de budget pour 2023, en hausse de 3,6 milliards d'euros par rapport à 2022, apporte une réponse lucide au problème du salaire des professeurs. Plus de 2 milliards d'euros financent des mesures de revalorisation des enseignants. d'abord, l'augmentation de 3,5 % de la valeur du point d'indice de la fonction publique bénéficie à plus d'un million de fonctionnaires dans le périmètre de la mission que nous examinons ce soir. soir. Surtout, la revalorisation des salaires, à hauteur de 10 % en moyenne, permettra de créer un choc d'attractivité du métier d'enseignant. On verra ! Vous le savez, dans sa lettre adressée à tous les enseignants le 16 septembre 2022, le Président de la République s'est engagé à ce qu'aucun qu'aucun professeur ne débute sa carrière en dessous de 2 000 euros net par mois à partir de la rentrée 2023. Cette mesure mobilisera 635 millions d'euros de crédits pour couvrir les mois de septembre à décembre 2023 et représentera 1,9 milliard d'euros en année pleine dès 2024. Enfin, une enveloppe additionnelle de 300 millions d'euros est prévue dans le projet de loi de finances pour 2023 afin d'apporter une rémunération complémentaire aux professeurs souhaitant prendre en charge missions supplémentaires. Par ailleurs, nous constatons que, malgré la diminution continue du nombre d'élèves due à la baisse des naissances en France, les effectifs des enseignants sont relativement stables. Il en résulte une hausse du taux d'encadrement des élèves, qui est non pas un hasard, mais bien le fruit d'un choix politique. Cette hausse résulte de la décision du Gouvernement de ne pas répercuter la totalité de cette baisse démographique sur l'emploi enseignant.

par la poursuite d'actions éducatives complémentaires aux enseignements, pour 188 millions d'euros. Je pense ici au dispositif « Devoirs faits

à l'enseignement technique agricole. Si celui-ci demeure une filière d'excellence, qu'il faut préserver, il est aussi un pilier de notre souveraineté alimentaire, dont la crise sanitaire a montré la grande importance. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera sans réserve les crédits de cette mission.